L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité

Monsieur le président, monsieur le président de la commission spéciale, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes réunis dans cet hémicycle pour examiner en première lecture le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité.

L’ensemble de ces initiatives contribuent à faire de la France une nation à la pointe de la cybersécurité. Il y a six semaines, je me présentais devant la commission spéciale constituée par votre assemblée pour examiner ce projet de loi.

désormais bel et bien d’un enjeu géopolitique. Je ne pouvais imaginer à quelle vitesse l’actualité nous rattraperait. Nous faisons face à une nouvelle réalité, qui s’impose à nous. Le 3 mars dernier, devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre exprimait sa préoccupation, face à une situation internationale qu’il décrivait comme « la plus grave, la plus déstabilisée et la plus dangereuse […] depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale surlendemain, dans son allocution relative au conflit en Ukraine, le Président de la République alertait quant à lui les Françaises et les Français face aux ingérences étrangères qui testent nos limites « dans les airs, en mer, dans l’espace et derrière nos écrans Nous sommes directement visés. Les tensions géologiques liées à la guerre en Ukraine, l’évolution des positions américaines ou encore le conflit au Proche Orient affectent directement notre sécurité numérique.

Pour autant, nous ne partons pas de zéro. Dès 2006, la France a fait le choix précurseur de mettre en œuvre un dispositif de protection des secteurs d’activité Dès 2016, à l’échelle de l’Union européenne, nous nous sommes dotés d’une première directive Network and Information Security, dite directive NIS 1, qui a établi les bases d’une sécurité renforcée pour les entités essentielles.

J’ai été particulièrement touchée par mes échanges avec les soignants de l’hôpital André Mignot, dans les Yvelines. Ces derniers sont encore marqués par les conséquences de la cyberattaque subie à vingt trois heures, le samedi 3 décembre 2022,

autant de situations contre lesquelles nous devons plus que jamais nous prémunir. Je tiens d’ailleurs à saluer devant vous la résilience et le sens du collectif dont font preuve les équipes que j’ai pu rencontrer. Qu’elles en soient sûres : l’État est à leurs côtés.

la France a joué un rôle précurseur dans la protection de ces infrastructures, avec le dispositif des secteurs d’activité d’importance vitale. Aujourd’hui, nous devons encore renforcer la capacité desdites entités à anticiper, à résister et à récupérer.

Parce que la menace n’a jamais été si diffuse, il était essentiel d’élargir le champ des entités couvertes. Nous avons conduit cette évolution en suivant quatre principes : concertation, proportionnalité, simplification et accompagnement. NIS 2 introduit une distinction claire entre deux types d’entités : d’une part, celles dites importantes, qui représentent 80 % des 15 000 entités couvertes, et pour lesquelles les obligations seront centrées sur une bonne hygiène numérique de l’autre, celles dites essentielles, qui seront soumises à des exigences de cybersécurité plus strictes et à des contrôles accrus, en amont comme en aval. Par ailleurs, nous avons fait le choix d’inclure 1 500 collectivités dans le C’est un choix assumé, qui s’explique avant tout par le fait que ces dernières sont la cible d’une attaque sur quatre recensée par l’Anssi, et ce dans tous nos territoires. J’assume tout autant de proposer que ces mêmes collectivités n’encourent pas de sanctions financières, puisqu’elles ne sont ni financées ni assurées dans les mêmes conditions qu’un organisme privé.

Les banques et les institutions financières sont toujours plus exposées au risque de cyberattaques. Selon le FMI, elles auraient subi plus de 20 000 incidents en vingt ans et connu une perte de 25 milliards d’euros entre 2020 et 2024.

Je souhaite m’assurer que cette transposition maintienne un niveau élevé de protection, sans compromettre la compétitivité de nos entreprises vis à vis de leurs concurrents, y compris européens.

d’abord, en rappelant que le coût d’une attaque cyber réussie est des dizaines de fois supérieur à celui de la mise en conformité et des mesures de protection ensuite, en indiquant que la rationalisation et l’harmonisation des pratiques de cybersécurité en Europe servent bien notre compétitivité, en évitant toute fragmentation réglementaire enfin, en soulignant que ce texte doit aussi permettre de supporter le développement de solutions technologiques nationales et européennes au sein d’un écosystème industriel innovant, créateur de valeur et d’emplois.

demandé à l’Anssi de travailler à un modèle de labellisation qui vous sera présenté dans le cadre des débats. Il permettra aux acteurs de faire valoir la résilience cyber non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité et un atout concurrentiel. enseignement est la nécessité, pour les entreprises et les collectivités, d’être guidées dans leurs nouvelles obligations. Je m’y attache, avec l’appui de l’Anssi, de la gendarmerie, de toutes les fédérations patronales et des associations.

à placer notre pays à la pointe du secteur stratégique de la cybersécurité. Ce texte doit aussi être l’occasion de sensibiliser largement le grand public La première des protections, c’est bien la pédagogie : nous devons tous, à notre niveau, contribuer à lever le tabou qui entoure encore bien trop souvent les cyberattaques. Je suis convaincue que les débats qui s’ouvrent seront constructifs et permettront d’aboutir à un texte simple et efficace, mais surtout utile à la sécurité des Françaises et des Français. La parole

Cette directive s’inspire en grande partie du dispositif français existant. Sa transposition en droit national consiste donc essentiellement en une actualisation du dispositif de sécurité des activités d’importance vitale, en vigueur depuis 2006 et désormais bien maîtrisé par les opérateurs concernés. Cette transposition marque toutefois un changement important de philosophie : elle acte le passage d’une logique de protection des infrastructures d’importance vitale à une approche axée sur la résilience. Cette orientation me semble pertinente, car il est évident que l’on ne pourra jamais se protéger contre toutes les menaces. L’enjeu est donc bien d’identifier les moyens d’assurer la continuité des activités essentielles pour le pays. qui concerne la transposition proprement dite, plusieurs différences doivent être signalées entre le texte qui nous est présenté et la directive. Les opérateurs exerçant dans le domaine de la défense ou de la sécurité nationale, qui étaient déjà soumis soumis au dispositif des SAIV, sont ainsi intégrés dans le champ de la transposition, alors que cela n’était pas prévu par la directive. Par ailleurs, la réalisation d’une analyse des dépendances à l’égard des tiers est prévue, une obligation qui ne figurait pas dans la directive REC. Enfin, les opérateurs d’importance vitale devront réaliser un plan de protection et de résilience pour chacun de leurs points d’importance vitale, comme c’est le cas dans le dispositif actuel, alors que la directive ne prévoit des plans qu’à l’échelle de l’opérateur lui même. Ces adaptations me semblent pertinentes au regard des objectifs du projet de loi. Par ailleurs, les autres obligations qu’il introduit – élaboration d’un plan de résilience opérateur, notification des incidents, instauration d’un mécanisme de sanctions administratives – sont conformes aux dispositions de la directive. À l’article 1, la commission spéciale a adopté plusieurs amendements visant notamment à définir les notions d’incident et de résilience, à préciser la date à partir de laquelle une astreinte prononcée dans le cadre d’une mise en demeure commence à s’appliquer, à fixer à vingt quatre heures le délai dans lequel l’opérateur doit signaler un incident à l’autorité administrative ou encore à renforcer les garanties d’indépendance de la commission des sanctions. Au sein du titre II, et notamment à l’article 6, la commission spéciale a adopté deux amendements visant à définir les notions d’incident et de vulnérabilité, qui ne sont pas présentes dans le projet de loi alors qu’elles figurent dans la directive NIS 2. Mes chers collègues, le dispositif de résilience des activités essentielles prévu par le présent projet de loi et amélioré par la commission spéciale renforcera notre capacité collective à faire face aux risques croissants. Cependant, beaucoup reste à faire, notamment quant à l’application concrète de ces dispositions et à leur déclinaison au niveau réglementaire. À ce titre, madame la ministre, nous veillerons particulièrement à ce que les services de l’État ne surtransposent pas la directive et accompagnent efficacement les opérateurs dans la mise en œuvre de ces nouvelles obligations. Il s’agit là d’une attente forte exprimée par les acteurs concernés.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en ma qualité de rapporteur chargé de l’examen du titre II du projet de loi, je centrerai mon intervention sur la transposition de la directive NIS 2. Comme nos auditions nous l’ont clairement montré, la menace cyber a largement changé de nature au cours des dix dernières années. Alors qu’elle ciblait avant tout les grandes entreprises, souvent à des fins d’espionnage industriel ou de déstabilisation, et était souvent d’origine étatique, elle est devenue systémique, émanant de plus en plus de groupes cybercriminels organisés, qui opèrent avant tout dans un but lucratif.

37 % de ces attaques visaient des TPE PME, 17 % des collectivités territoriales, 4 % des établissements de santé et 12 % des établissements d’enseignement supérieur. Les conséquences de ces attaques peuvent être particulièrement pénalisantes pour les entités, ainsi que pour leurs usagers ou leurs clients, voire provoquer des faillites ou mettre des vies en danger.

Le premier est de faire entrer dans le champ des entités régulées les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communautés de communes et les communes de plus de 30 000 habitants.

nombre des amendements adoptés par la commission spéciale ont visé à répondre au constat d’une « sous transposition », qui laissait une place trop importante aux dispositions de nature réglementaire. ses amendements, la commission spéciale a beaucoup insisté également sur la nécessaire proportionnalité des mesures de cybersécurité qui seront imposées, par un référentiel de l’Anssi, aux entités régulées. Il convient de tenir compte systématiquement de la taille de l’entité, du degré de son exposition aux risques cyber, de la probabilité de survenance d’incidents et de leur gravité, afin de ne pas imposer des obligations excessives et trop coûteuses.

pour faire connaître et faire comprendre les nouvelles obligations prévues par la réglementation, et assurer leur mise en œuvre effective. Il faudra donc également ne pas prévoir de contrôle ni,, de sanctions pendant la période de montée en puissance cyber. La parole

qui prévoit que la politique de gestion des risques liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC) des secteurs bancaire, assurantiel et financier est conforme au règlement Dora du 14 décembre 2022. Le paquet Dora constitue la déclinaison de la directive NIS 2 applicable au secteur financier, qui est en effet une cible de choix pour les cyberattaques. Le niveau élevé d’interconnexion du secteur constitue

Les menaces cyber, en forte augmentation depuis plusieurs années, représentent ainsi, selon la Banque de France, un risque très élevé, supérieur au risque de marché et au risque climatique.

en fusionnant les dispositifs de déclaration d’incidents opérationnels ou de sécurité liés au paiement, prévus par la directive sur les services de paiement, et le dispositif de déclaration d’incidents liés aux TIC, prévu par le règlement Dora ; à l’article 43 en créant un guichet unique, permettant au passage à la France de respecter l’article 19 du règlement Dora, qui impose, lorsque c’est nécessaire, de désigner une seule autorité compétente pour la notification des incidents. Je vous proposerai d’ailleurs un amendement visant à instituer l’Autorité des marchés financiers comme guichet unique pour les entreprises de marché et pour les prestataires de services sur cryptoactifs.

au début du mois, le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a ordonné la suspension des opérations cyber concernant la Russie. Cette démarche participe du processus de rapprochement mené par l’administration Trump. Afin de conclure une paix factice, c’est à dire de concéder la victoire à Poutine, les États Unis sont en train de redonner des marges de manœuvre à la Russie, même si des revirements semblent se profiler à l’occasion des discussions en cours en Arabie saoudite qui, espérons le, aboutiront à une solution favorable. fait, depuis la nouvelle invasion russe de l’Ukraine le 24 février 2022, une guerre de haute intensité est menée sur notre continent. Offensives et contre offensives, guerre de tranchées, guerre des drones, tous les moyens sont employés dans cette lutte. lutte. Or, à l’heure de la trahison de Trump, force est de constater, à regret, que les troupes russes avancent plus rapidement. Si 2 000 kilomètres nous séparent de Kiev, ce serait une erreur de conclure que ce conflit ne nous concerne pas directement des sabotages ont lieu partout en Europe et les opérations dans le champ informationnel – faux cercueils recouverts de drapeaux français près de la tour Eiffel, étoiles de David

Sans l’avoir déclarée et en prenant bien soin de rester sous le seuil de la conflictualité ouverte, la Russie mène une guerre contre notre pays, contre nos intérêts, jusque sur notre territoire. Dans son combat, le Kremlin encourage la pègre à mener contre nous des attaques cyber, lorsqu’il ne les lance pas lui même. Il y a un an, jour pour jour, c’est le réseau interministériel de l’État qui était visé, et les différents ministères avaient

La France et ses partenaires européens doivent réagir pour défendre efficacement leurs concitoyens. Plusieurs directives européennes – REC, NIS 2, Dora – ont ainsi été adoptées pour identifier plus clairement les infrastructures et services essentiels au bon fonctionnement de nos sociétés.

Le texte que nous examinons prévoit des sanctions en cas de violation de ses dispositions. Sans doute seront elles rares, puisque tous les acteurs concernés ont un intérêt direct à assurer leur propre sécurité. Elles sont néanmoins indispensables pour protéger nos concitoyens tant contre la négligence fautive que contre la malveillance caractérisée. Ce texte technique ne fera sans doute pas la une des journaux. Il est pourtant, mes chers collègues, d’une importance capitale. De sa bonne mise en œuvre dépendent la sauvegarde de notre activité économique et,, la sécurité de nos entreprises, de nos collectivités territoriales, de nos services publics et de nos concitoyens. Ce cadre devra bien entendu s’adapter aux évolutions technologiques et être réévalué assez régulièrement pour rester pertinent. Avant de conclure, je voudrais réaffirmer que la réglementation ne suffira pas. sécurité implique la souveraineté. La plupart des infrastructures et outils numériques que nous utilisons sont conçus aux États Unis et fabriqués en Chine. C’était déjà problématique avant la deuxième présidence Trump ; cela devient extrêmement critique.

songe aux antennes 5G, voire aux grues chinoises employées dans les ports américains ! Rappelons que Washington avait alerté sur la vulnérabilité des matériels et logiciels qui sont conçus par des puissances hostiles. À l’heure où les Européens n’ont plus d’autres vrais amis qu’eux mêmes, il est grand temps

L’industrie européenne devra bien sûr respecter une logique de rentabilité, mais aussi intégrer le fait que la souveraineté, comme la liberté – notre liberté chérie –, a un prix qui mérite d’être payé. La parole

trois directives européennes, représente indéniablement une avancée majeure pour la protection de notre pays face aux menaces actuelles. Nous devons saisir cette occasion pour devons saisir cette occasion pour aller encore plus loin, en particulier en matière de sécurité de nos infrastructures numériques, devenues indispensables à notre vie quotidienne, à notre économie et à la continuité même des services essentiels de la Nation. de la Nation. J’attire votre attention sur un point crucial : la reconnaissance et la protection renforcée des infrastructures des réseaux de communications électroniques et, plus spécifiquement, de la fibre optique et des antennes relais de téléphonie mobile. Il serait utile de clarifier leur statut au sein même du code de la défense. En effet, il nous faudrait reconnaître explicitement ces infrastructures comme des activités numériques Cette classification serait loin d’être symbolique. Elle entraînerait l’application d’obligations de sécurité renforcée pour les opérateurs, à la hauteur des enjeux stratégiques qu’elles représentent. Il serait également utile de ne pas les considérer comme un bloc monolithique. Nous devrions ainsi distinguer les différents types d’infrastructures de fibre optique et de téléphonie mobile en fonction de leur criticité et de leur impact potentiel sur les citoyens en cas de défaillance ou d’attaque. Une simple armoire de rue n’a évidemment pas le même niveau de criticité stratégique qu’un nœud de raccordement optique, un central téléphonique ou un pylône d’antenne relais. Aborder ces aspects dans la loi impliquerait également la définition d’exigences de sécurité qui soient véritablement spécifiques et adaptées à ces infrastructures numériques vitales, autour de trois dimensions de la sécurité la sécurité physique, modulée en fonction de la criticité des équipements ; la sécurité logique, pour protéger les systèmes d’information associés à ces infrastructures et garantir la mise en œuvre de plans de continuité et de reprise d’activité robustes ; la sécurité environnementale, trop souvent négligée, pour assurer la protection de ces infrastructures face aux aléas extérieurs. Enfin, il faudrait renforcer et surtout clarifier les obligations qui pèsent sur les opérateurs exploitant ces activités d’importance vitale numériques. Là encore, il me semble essentiel de les préciser dans la loi, pour que ces exigences de sécurité spécifiques ne restent pas lettre morte. Mes chers collègues, la tempête Alex, qui a frappé si durement les Alpes Maritimes en 2020, n’est pas un cas isolé. Je peux témoigner, pour l’avoir vécue, de la vulnérabilité de nos infrastructures numériques.

isolement. Elle a démontré de façon brutale l’importance cruciale de renforcer la résilience de ces infrastructures face aux aléas climatiques, mais aussi aux actes de malveillance, afin de garantir, en toutes circonstances, la continuité des services essentiels pour nos concitoyens. Les exigences nouvelles en matière de cybersécurité transposées dans ce projet de loi font écho à la résilience et à la robustesse des réseaux de communication. Et si l’on convient qu’elles sont indispensables, elles représentent par ailleurs un défi significatif, en particulier pour nos collectivités territoriales. La transposition de la directive NIS 2 étend ces obligations à un grand nombre d’établissements publics de coopération intercommunale, notamment aux plus petites intercommunalités à fiscalité propre, comme les communautés de communes. Or ces structures ne disposent pas toujours des moyens humains, financiers ou de l’ingénierie nécessaires pour se mettre en conformité avec ces nouvelles L’expérience du plan France Relance et de son parcours cybersécurité a démontré l’importance d’un accompagnement ciblé. Toutefois, force est de constater que ce dispositif n’a bénéficié qu’à une minorité de petites intercommunalités.

La France, comme le reste du monde, est confrontée à une menace croissante dans le domaine du numérique. Dans un contexte géopolitique et sécuritaire dégradé, les infrastructures les plus critiques, déjà soumises aux risques naturels et technologiques, peuvent être régulièrement ciblées par des actions malveillantes. Ces actions visent tant les installations physiques que leurs systèmes d’information. Selon Statista, un tiers des Français a déjà été victime d’une cyberattaque et les trois quarts des entreprises françaises ont subi au moins une attaque de type cyber en 2024. Ces attaques ne se limitent pas aux personnes et aux entreprises privées. Réseaux hospitaliers, collectivités territoriales, intranet de nos écoles ou encore sites internet institutionnels sont tout autant des cibles vulnérables pour des personnes malveillantes. Les infrastructures critiques de notre pays, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports ou de la santé, subissent ainsi une menace constante. Les Les enjeux sont très importants. Une perturbation de ces infrastructures pourrait, et peut déjà actuellement, avoir des conséquences désastreuses sur la sécurité nationale, l’économie de notre pays ou la santé de nos concitoyens. Face à cette menace croissante, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui vise à mieux nous prémunir contre ce danger nouveau. Il vise ainsi à renforcer la résilience de nos infrastructures critiques et à améliorer notre cybersécurité en transposant dans notre droit national trois directives trois directives européennes. La directive sur la résilience des entités critiques tend à renforcer la capacité de ces acteurs à résister aux perturbations naturelles et humaines. En transposant cette première directive, le projet de loi permettra de renforcer la résilience de nos infrastructures par l’élargissement du nombre de secteurs concernés, par une meilleure prise en compte des interdépendances des interdépendances entre ces secteurs, y compris entre États membres, ou encore par une obligation de notification des incidents majeurs. Les opérateurs de ces infrastructures devront ainsi adopter des mesures spécifiques pour assurer la continuité de leurs services en cas de perturbation. Ce texte prévoit en effet le passage d’une logique de protection physique des infrastructures à une logique de résilience et de continuité d’activité. La directive NIS 2 établit, quant à elle, des exigences de cybersécurité pour les entités de secteurs essentiels.

s’enregistrer auprès d’une autorité nationale, notifier les incidents importants à cette autorité et mettre en œuvre des mesures adaptées de gestion des risques en la matière. Enfin, la directive Dora, également transcrite dans ce texte, a pour objet de garantir que le secteur financier puisse continuer à fonctionner même en cas de perturbation majeure, en renforçant, à la fois, la protection des données des clients et le rôle des autorités de de surveillance, tout en établissant des règles équitables dans l’Union européenne. Ces trois directives et l’ensemble des mesures qu’elles contiennent constituent une réponse coordonnée au niveau européen pour faire face aux menaces croissantes pesant sur nos infrastructures critiques et notre cybersécurité.

dispenser les collectivités des sanctions pécuniaires prévues en cas de manquement aux obligations de sécurité des systèmes d’information. Mes chers collègues, il est inutile de vous rappeler les méthodes employées par certains États, notamment la Russie, afin de déstabiliser des pays européens et influer sur leurs décisions et processus démocratiques. Face à des cybermenaces de plus en plus sophistiquées, globalisées et émanant des quatre coins du monde, il est primordial que nous ne fassions plus preuve de naïveté sur ces questions, et que nous puissions coordonner notre réponse avec nos alliés européens. Dans la lutte contre la menace cyber, le rôle de l’État doit être central. Il y va de la confiance de nos entreprises et de nos concitoyens, qui doivent être protégés par un État fort et souverain,

Cependant, lorsque le progrès avance, de nouvelles menaces font leur apparition. Il faut ainsi choisir entre les subir ou s’en prémunir. Il est de notre devoir de nous adapter de nous adapter à ce défi, auquel ce projet de loi apporte une réponse ambitieuse et nécessaire grâce à l’adaptation de notre législation au droit européen. Aussi, le groupe RDPI votera ce texte.

Corbeil Essonnes, Villefranche sur Saône, Dax, Charleville Mézières, Arles, Cannes : voilà une liste non exhaustive de communes dont les hôpitaux ont été la cible de cyberattaques ces dernières années. Comme le souligne régulièrement l’Anssi, les cybercriminels ciblent de plus en plus régulièrement, sur le territoire français, des hôpitaux à l’aide de rançongiciels, paralysant ainsi l’activité de structures vitales de l’État. Les conséquences de ces cyberattaques sont évidemment dramatiques. Elles déstabilisent profondément et parfois durablement le fonctionnement des établissements qui en sont victimes. Elles constituent une grave violation du droit à la vie privée, les données volées pouvant être vendues à des tiers, ou encore être utilisées à des fins d’usurpation d’identité.

Elle impose une application uniforme des obligations de sécurité et de continuité des activités, afin de doter l’ensemble des opérateurs du marché intérieur de standards de sécurité communs, tout en préservant la concurrence. ce projet de loi est également, en plus de sécuriser les 500 infrastructures critiques, d’assurer la résilience de 15 000 entités dites « essentielles » ou « importantes » et de l’ensemble de leurs systèmes d’information, afin de faire face au risque de cyberattaques, qu’il s’agisse d’hameçonnage, de rançongiciel ou d’exploitation de diverses vulnérabilités des systèmes. Enfin, le texte renforce la résilience opérationnelle du secteur financier européen en matière de cybersécurité et de gestion des risques informatiques. informatiques. Les entités financières auront l’obligation de mettre en place des cadres complets de gouvernance des risques liés aux technologies de l’information et de la communication, et de respecter des normes strictes de protection des données des clients. Il est prévu que l’Anssi, dans sa fonction de contrôle, puisse prononcer des sanctions administratives et financières, d’un montant allant jusqu’à 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires, et imposer une procédure de mise en conformité. Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics administratifs sont visés par ce texte. des sanctions financières, parfois lourdes, en cas de manquement ne paraît pas adapté à leur situation, alors qu’elles font déjà face à des contraintes financières croissantes. La réalité est que 73 % des petites et moyennes collectivités ne peuvent se permettre de consacrer plus de 5 000 euros par an à l’informatique et à la sécurité des systèmes. Européen a déposé plusieurs amendements visant à prendre en compte l’impératif donné aux collectivités de maîtriser leurs dépenses dans un contexte de baisse de leurs ressources financières. Nous proposons de les exonérer de sanctions financières en cas de manquement aux obligations de sécurisation des systèmes d’information. Nous appelons à privilégier des approches alternatives, telles que l’accompagnement, la formation et le soutien technique. Le groupe du RDSE a également déposé un amendement réduisant l’astreinte pouvant être appliquée à une collectivité de 5 000 euros à 100 euros par jour. Nous proposons aussi d’exonérer du financement des audits les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics administratifs. L’imposition d’un contrôle à leur charge représenterait une contrainte financière supplémentaire, qui risquerait d’entraver leur fonctionnement et de compromettre leur équilibre budgétaire. Enfin, il nous semble raisonnable de laisser un délai de cinq ans pour appliquer les nouvelles règles, ce qui permettrait à l’État d’accompagner les collectivités territoriales dans leur mise en œuvre, par une évaluation des moyens et par la mise en place d’une offre de formation. Ce texte est nécessaire, mais les obstacles sont multiples. De nombreuses PME sont limitées par des questions de trésorerie : les solutions de détection ne sont pas toujours à leur portée ; elles manquent parfois de ressources humaines ou d’une connaissance des réglementations. Nous devons veiller à ce que les obligations adoptées soient proportionnées à la situation de l’entité concernée, et à ce que les collectivités, qui sont en première ligne dans la lutte contre les menaces cyber, bénéficient d’un accompagnement de l’État tout au long du processus.

Je souscris en tout point aux constats et aux observations des rapporteurs Michel Canévet, Patrick Chaize et Hugues Saury, qui ont fait évoluer le texte dans le bon sens –

ainsi que celui de nos collègues qui ont largement participé aux travaux de la commission spéciale et contribué à l’élaboration du texte par leurs amendements, souvent inspirés par les auditions des représentants de l’écosystème.

Ce texte était très attendu par l’ensemble des professionnels et des parties prenantes des secteurs privé et public, car la transposition de la directive NIS 2 devait intervenir avant le 17 octobre 2024.

dans le domaine de la cybersécurité, un effort tout particulier en matière de sensibilisation et de prise en compte de la gravité des risques encourus. Je participe à cet effort en tant que rapporteur sur les crédits de l’Anssi depuis 2017. En 2023, les cyberattaques ont coûté près de 90 milliards d’euros à l’économie française.

Notre devoir est de faire prendre conscience à nos concitoyens des menaces cyber qui pèsent sur eux. Notre objectif premier n’est pas d’empêcher les cyberattaques. Elles ne pourront que s’accentuer dans les années qui viennent – c’est un fait. Vous avez indiqué, madame la ministre, que la

Je voudrais ici relayer quelques unes des nombreuses observations qui nous ont été faites. J’ai relevé un premier paradoxe. Bien que l’Anssi ait indiqué avoir conduit, depuis septembre 2023, des consultations avec plus de soixante dix fédérations professionnelles,

Cela soulève un second paradoxe. De nombreux intervenants ont souligné l’absence de transposition de certaines dispositions figurant dans les directives, telles que les définitions des notions de périmètre d’activité, d’incidents et de délais.

De fait, ni les acteurs concernés ni la commission spéciale n’ont été rassurés sur la méthode de concertation et d’élaboration de ces derniers. J’ai eu plusieurs fois le sentiment que le projet de loi donnait carte blanche à l’administration, sans que le législateur ait son mot à dire. C’est pourquoi la commission spéciale a formulé plusieurs recommandations à l’attention du Gouvernement : premièrement, veiller à la proportionnalité des obligations des entités assujetties ; deuxièmement, fournir un effort de simplification des mesures d’application se garder de toute surtransposition réglementaire ; quatrièmement, enfin, accompagner les collectivités territoriales dans cette démarche nouvelle, en tenant compte des problématiques de compétences et de financement. À titre plus personnel, j’estime, avec mon groupe, qu’il est important que le projet de loi ne soit pas perçu comme un catalogue inintelligible d’obligations et de sanctions. Il doit au contraire faire valoir une vision positive de l’élévation du niveau de résilience et de cybersécurité de tout le pays. Plus largement, et pour conclure en ce qui concerne la dimension européenne de cette transposition, je voudrais poser la question de l’harmonisation européenne, ou plutôt, devrais je dire, du risque de non harmonisation, source de distorsions de concurrence avec nos voisins européens. Un exemple précis vaut mieux qu’un long discours : comme l’a rappelé opportunément notre collègue Vanina Paoli Gagin, nos voisins belges ont déjà transposé la directive NIS 2.

clairement de trouver le point d’équilibre entre le besoin légitime de sécurité nationale et l’acceptation des normes par les acteurs concernés. Ce processus ne peut être laissé à la seule discrétion d’une agence qui ne rend aucun compte devant les entreprises et les collectivités. J’en appelle à vous, madame la ministre, pour élever

ne soit pas possible d’imposer aux fournisseurs de services de chiffrement d’intégrer des dispositifs techniques visant à affaiblir volontairement la sécurité de leurs systèmes. Garantir la sécurité numérique constitue un véritable enjeu du texte. Laisser des brèches dans le cryptage des données, des « portes dérobées », appelées, peut poser de véritables problèmes. Fragiliser la sécurité des solutions de chiffrement françaises et européennes nuirait à notre compétitivité face aux acteurs internationaux. Cet amendement a reçu de nombreux soutiens de la part des acteurs du numérique. Votre avis, madame la ministre, fera l’objet Je vous inviterai, mes chers collègues, à voter mon amendement. Notre travail ne sera pas terminé avec le vote du texte. Pour être efficace, le projet de loi doit être largement accepté par tous. Cela dépendra de la qualité du dispositif qui sera retenu

Le monde s’embrase ; nous assistons à une militarisation croissante d’internet et à une explosion de la cybercriminalité. En ce sens, la cybersécurité s’impose aujourd’hui comme un enjeu stratégique, qui irrigue l’ensemble des sphères de notre société, de nos institutions et de notre économie. Si le texte dont nous débattons aujourd’hui répond à certaines urgences, il demeure en deçà des véritables enjeux. Il est, en réalité, le produit d’une doctrine politique qui s’est résignée à la dépendance, préférant la résilience à la souveraineté, l’adaptation à la maîtrise, la soumission aux rapports de force du capitalisme numérique mondialisé plutôt que la reconquête de nos capacités industrielles et technologiques. Alors que la France était le pays de référence en matière de savoir faire et de conception de produits numériques à grande échelle, notre dépendance technologique n’a jamais été aussi grande vis à vis du et des logiciels américains. Pourtant, comme le soulignent de nombreux chercheurs, nous avons été capables de déployer intégralement des réseaux filaires,

d’un tissu industriel et de recherche national. Mais les gouvernements successifs ont fait le choix de la désindustrialisation dans les secteurs des télécoms et de l’électronique grand public.

Ommic, fleuron français de semi conducteurs pour l’industrie des télécommunications et le domaine spatial, a lui aussi été vendu. De nos jours, le Gouvernement continue de délaisser Atos. La privatisation et l’ouverture à la concurrence des réseaux téléphoniques ont balayé les laboratoires de recherche de France Télécom. Les résultats de ces renoncements sont criants

et captent la valeur de notre propre développement numérique. À l’heure actuelle, la France importe près de 20 milliards d’euros de technologies chaque année. Loin d’être un acteur de la révolution numérique en cours, nous en sommes devenus les consommateurs passifs, tributaires des infrastructures étrangères, prisonniers de systèmes d’exploitation, de solutions logicielles et de services extraterritoriaux. Nous n’embrassons pas le futur, nous l’achetons ou nous le louons ! Le texte dont nous débattons aujourd’hui est le résultat de cet abandon d’une volonté de souveraineté numérique. Cette dernière laisse la place à la notion de résilience. En effet, cette notion, centrale dans ce nouveau train de directives, traduit une stratégie orientée vers l’aval de la chaîne de valeur, sécurisation des solutions logicielles, des architectures réseau et des systèmes d’information, de nouvelles obligations de et la surveillance des prestataires de technologies critiques.

Au delà des coûts, c’est la possibilité même de trouver des personnels suffisamment qualifiés pour mettre en œuvre ces dispositions qui suscite des interrogations dans certaines régions où les ressources humaines sont rares et où, nous le savons, le recours aux prestataires de cybersécurité se traduira par des hausses de prix, dont les conséquences financières sont mal anticipées par le Gouvernement. cette interrogation sur les compétences est l’aboutissement de choix politiques d’externalisation des compétences et de plateformisation de l’action publique. Ce texte, malheureusement, ne permettra pas d’enrayer la concentration des ressources et des services critiques entre les mains de grandes entreprises transnationales, majoritairement extraeuropéennes – IBM, Intel, Google, Microsoft, Amazon, etc. Or cela conditionne directement l’autonomie stratégique des États et leur capacité à définir les futurs modèles de production et d’innovation industrielles.

C’est dans ce contexte que nous devons adapter notre droit et nous prononcer sur le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, lequel transpose trois directives européennes : Dora, REC et NIS 2. Celles ci nous permettront de protéger nos collectivités, nos infrastructures critiques et nos entreprises face à la cybercriminalité.

notamment à la santé publique et à l’environnement. Par ailleurs, la définition des infrastructures critiques retenue dans le projet de loi permet d’aller plus loin que ce qui est prévu dans la directive,

à un accroissement général de la cybermenace. Nos infrastructures critiques sont déjà concernées par ces enjeux. Désormais, nos collectivités sont aussi vulnérables face à ce risque. Les récentes attaques contre nos mairies ou nos hôpitaux nous rappellent qu’il est nécessaire d’anticiper la menace.

Si le groupe écologiste salue cette volonté de mettre en œuvre une véritable protection et d’assurer la résilience de nos infrastructures critiques et de nos collectivités, il émet néanmoins quelques réserves sur les moyens dont disposent l’ensemble des acteurs concernés tant dans la mise en œuvre des dispositions de NIS 2

par an pour les collectivités, alors même que nombre d’entre elles manquent de ressources humaines et techniques en cybersécurité. Nous regrettons ainsi l’absence d’un véritable plan d’accompagnement des acteurs, qui aurait permis de conforter l’approche visant à renforcer nous déplorons l’instauration de sanctions financières importantes, dans un contexte où les collectivités, leurs groupements et leurs établissements publics administratifs souffrent d’ores et déjà de fortes contraintes budgétaires. Imposer des sanctions financières à ces entités pourrait aggraver leur situation budgétaire déjà précaire, comme en témoignent les récentes inquiétudes exprimées par les élus départementaux face aux contraintes financières croissantes. Aussi, le groupe écologiste proposera par voie d’amendement une exonération des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs des sanctions financières prévues en cas de manquement aux obligations de sécurité des systèmes d’information, afin d’éviter des contraintes supplémentaires. Nous aurions aimé qu’une approche alternative aux sanctions financières soit mise en place autour d’un véritable plan national d’accompagnement. Cela aurait permis de clarifier le rôle des centres que les modalités de l’accompagnement de ces entités nouvellement soumises à la directive NIS2 et de la mutualisation des moyens de nos collectivités. Mes chers collègues, nous le savons, ce projet de loi est nécessaire. Il permet des avancées en apportant des réponses aux enjeux vitaux de la cybersécurité et en amorçant la réflexion sur la construction d’une cybersécurité cybersécurité territoriale. Néanmoins, les circonstances budgétaires ne permettent pas aux acteurs concernés d’avancer dans cette voie sereinement. Une approche solidaire d’accompagnement par l’État est essentielle pour éviter que les petites collectivités ne soient laissées seules face aux cybermenaces. Celles ci sont en progression sur notre sol et ne peuvent nous laisser sans réaction. C’est pourquoi le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera pour ce projet de loi, même si nous aurions souhaité aller plus loin dans l’élaboration d’une stratégie européenne de nature à nous assurer autonomie et souveraineté en la matière. La parole

du 1 au 3 avril 2025, Lille accueillera, comme chaque année, le Forum international de la cybersécurité (FIC), qui réunit les principaux acteurs du secteur. C’est dire si l’enjeu cyber est bien identifié dans cette ville. Et pourtant, en mars 2023, elle a subi une intrusion dans son système informatique dont le coût a été évalué à près de 2 millions d’euros. Certes, les assurances couvriront une partie des frais et aucune donnée n’a été perdue, mais le fonctionnement habituel de la collectivité a été fortement perturbé. Lille a été victime d’une attaque malgré l’écosystème cyber qui l’entoure. Une collectivité sur dix déclare l’avoir été dans les douze derniers mois, d’après le baromètre de la

Une législation européenne en construction permanente tente de faire face à ces évolutions technologiques rapides et de contrer les attaques d’ampleur par une meilleure prévention et une plus grande coordination entre les États membres. Comme nous l’avions signalé dans la proposition de résolution européenne présentée avec Catherine Morin Desailly et Cyril Pellevat, il faut prendre garde à ce que cet enchaînement de textes européens ne complexifie pas l’ensemble du paysage en matière de cybersécurité. Nous devons aussi veiller au financement de tous les investissements induits. Cette question financière est l’une de celles qui se posent dans le cadre du projet de loi que nous examinons et qui a pour objet de transposer – enfin, oserai je dire la directive sur la résilience des entités critiques, la directive NIS 2, qui étend le dispositif actuel de prévention et de protection à un plus large tissu économique et social ainsi qu’au secteur public, et le règlement Dora, applicable aux entités financières. Avec ces textes, c’est un changement d’échelle qui s’opère en ce qui concerne tant les exigences de sécurisation des systèmes d’information et de résilience que les catégories d’entités visées.

publiques et privées est de taille : il importe de mieux se protéger, comme le montre mon exemple lillois. Cependant, le retard collectif d’investissement dans le domaine de la cybersécurité ne sera pas aisé à rattraper. Les fortes tensions sur la filière des métiers cyber nous semblent être un point d’alerte majeur, tout comme les coûts en matière d’infrastructures, de formation et de mise en conformité, qui peuvent être lourds à supporter pour toutes les entités.

La plupart des amendements du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain visent donc à assurer une montée en puissance réellement progressive et faisant l’objet d’une concertation régulière de la future loi, avec un accompagnement opérationnel et financier qui tienne mieux compte des capacités de chacun. C’est pour nous la condition de l’acceptabilité du projet de loi. pas de date d’application, mais il comporte des contrôles et des sanctions. Or l’enjeu cyber ne peut pas être vécu comme punitif. Rançongiciel, hameçonnage, déni de service : oui, la menace est réelle ; oui, nous avons besoin d’une meilleure cyberprotection, mais rien ne serait pire que des blocages dans les esprits et sur le terrain, parce qu’on oblige et on sanctionne au lieu d’expliquer et d’aider. Le rôle de l’Anssi est à cet égard précieux, mais elle ne pourra pas tout faire, tout de suite et toute seule. Aussi, dans le droit fil des travaux de la commission spéciale et des ajouts qui ont nous souhaitons vivement que la stratégie nationale cyber suggérée par le rapporteur Patrick Chaize soit complétée par des éléments concrets et territoriaux, comme un plan d’accompagnement local ou un sous préfet chargé de ces

par nos collègues Rémi Cardon et Sébastien Meurant dans leur rapport sur la cybersécurité des entreprises. Face aux cybermenaces croissantes issues de groupes criminels privés

de loi. Ce texte de loi transcrit en droit français trois directives européennes essentielles pour adapter notre cadre juridique à cette menace croissante. La première est la directive REC, qui modernise notre approche en passant d’une logique de protection à une véritable stratégie de résilience des infrastructures critiques.

Ce projet de loi est essentiel au regard de la montée en puissance des cyberattaques, et notamment des rançongiciels. C’est une menace qui touche toutes nos infrastructures vitales. Établissements stratégiques, hôpitaux, collectivités locales, et même petites et moyennes entreprises : personne n’est à l’abri Comme le rappellent Patrick Chaize, Hugues Saury et Michel Canévet dans leur rapport, en un an, les attaques ont bondi de 30 %, avec des conséquences économiques et sociales considérables.

Je forme donc le vœu que l’examen en séance publique suive une dynamique similaire. Pour autant, aussi nécessaire soit il, ce texte soulève encore des questions et appelle des engagements clairs du Gouvernement. J’espère que le débat de ce soir permettra d’apporter des réponses. La mise en œuvre des obligations ainsi transposées risque de peser sur les collectivités territoriales et les entreprises, en particulier sur les plus petites d’entre elles. Au niveau réglementaire, un cadre clair et réaliste doit être défini pour éviter toute surtransposition excessive. Un accompagnement financier et technique sera indispensable pour que les entités concernées puissent réellement se conformer aux exigences de cybersécurité. Je n’oublie pas la question de la coordination et du contrôle, à laquelle il faudra apporter des réponses réalistes et pragmatiques.

ailleurs, quelle sera la place laissée à l’harmonisation européenne afin d’éviter des doublons et des contraintes disproportionnées pour nos entreprises ? Enfin, l’examen du texte devra permettre de clarifier et de renforcer certains points essentiels, comme les seuils de classification des entités essentielles et importantes ou encore l’accompagnement des acteurs privés et publics, lequel doit être renforcé pour garantir une application efficace et proportionnée des obligations de cybersécurité. Nous devons légiférer vite, car le temps nous est compté et la transposition de certaines dispositions est déjà en retard. C’est le cas notamment de NIS 2. Pour autant, ne confondons pas vitesse et précipitation. Ce texte est un premier pas indispensable, mais sa réussite dépendra des mesures concrètes d’accompagnement et de mise en œuvre que le Gouvernement devra impérativement détailler.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il est sept heures du matin, quelque part en France, lorsqu’un dysfonctionnement touche une station de traitement d’eau potable desservant une métropole de plusieurs centaines de milliers d’habitants. Du fait du manque d’anticipation, le service n’est pas rétabli aussitôt, et ce qui est d’abord un incident isolé devient une panne qui s’aggrave en quelques heures : les réservoirs se vident et le réseau de distribution cesse de fonctionner. Dans les hôpitaux, dans les industries, on rationne la consommation ; la population panique et les autorités peinent à coordonner la réponse d’urgence. Et le pire, c’est que ce n’est ni une attaque ni une catastrophe naturelle qui est la cause de tout cela, mais une simple défaillance technique aggravée par un manque de planification, d’anticipation et de résilience. Cette situation est techniquement parfaitement vraisemblable. Il est des textes qui surgissent dans nos débats parlementaires comme une évidence au vu du contexte que nous traversons. Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui appartient à cette catégorie. Regardons au delà de la France, comme l’ont fait quelques uns des orateurs précédents. Le tragique de l’Histoire, imposé à l’Ukraine depuis trois ans, a mis en évidence la vulnérabilité des infrastructures critiques déjà soumises aux risques naturels et aux attaques physiques et cyber, qui se sont intensifiées ces dernières années. À cet égard, la transposition de la directive REC dans le titre I du présent projet de loi, sur lequel je concentrerai mon intervention, ne fait que tirer les conséquences d’une réalité incontestable : la vulnérabilité croissante de nos infrastructures essentielles dans un monde où les crises deviennent la norme. Nous avons ainsi vécu une crise sanitaire qui a révélé les fragilités de nos chaînes logistiques. Nous avons vu ces dernières années des collectivités tétanisées par des cyberattaques, des entreprises stratégiques paralysées par des rançongiciels, des États étrangers déployer leur influence par la manipulation de l’information et le sabotage économique. Nos infrastructures critiques sont non plus simplement des rouages invisibles de notre quotidien, mais des cibles, des vulnérabilités, des enjeux de puissance. Les yeux des gouvernants se dessillent enfin face aux menaces des impérialismes russes et chinois, mais aussi américains.

mais il utilise la transposition pour réviser cette politique publique essentielle. Il acte une évolution conceptuelle importante : nous sommes non plus dans une logique de protection statique des infrastructures, mais dans une approche dynamique de résilience. Cette réforme normative constitue ainsi l’opportunité de moderniser notre organisation nationale : rationalisation de la classification du dispositif, simplification des documents de planification requis ou encore renforcement des modalités de supervision. égard, la multiplication par cinq du nombre d’opérateurs d’importance vitale, qui passera de 300 à près de 1 500, est révélatrice de la nécessité d’une vigilance accrue, dans un monde où les risques sont de plus en plus systémiques et interdépendants.

Belrhiti. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous étudions aujourd’hui revêt une importance capitale : la protection et la résilience de nos infrastructures critiques face au renforcement au renforcement des cyberattaques. Dans un monde où les menaces numériques se multiplient et où nos infrastructures essentielles interconnectées sont de plus en plus exposées au risque cyber, nous avons le devoir de doter notre pays des outils nécessaires pour protéger ses intérêts fondamentaux. Ce texte, qui transpose notamment les directives européennes NIS 2 et REC, constitue une avancée majeure dans ce domaine, mais il exige de notre part une vigilance accrue et un engagement sans faille. Il ne se passe plus une semaine sans que des cyberattaques viennent nous rappeler la vulnérabilité de nos infrastructures numériques. Rappelons que les attaquants se saisissent de toutes les faiblesses techniques de nos systèmes d’information. Des hôpitaux ont été paralysés, des collectivités territoriales prises en otage par des rançongiciels et des entreprises clés de notre économie et de notre base industrielle et (BITD) ciblées par des actes de cyberespionnage. La liste est longue et les conséquences sont désastreuses. La France subit une pression constante et omniprésente dans le cyberespace. En 2024, les événements de sécurité portés à la connaissance de l’Anssi ont connu une augmentation de 15

les compétences des acteurs désignés, mais également de souligner ses diverses faiblesses, lesquelles ont depuis été corrigées. Ainsi, le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité vise à répondre à ces défis en transposant plusieurs directives européennes qui s’articuleront correctement avec notre législation nationale. Il prévoit notamment une meilleure identification des entités essentielles et importantes, une responsabilisation accrue des dirigeants en matière de cybersécurité et des sanctions plus dissuasives en cas de manquement pour les opérateurs négligents. S’il constitue une avancée significative, sa mise en œuvre nécessitera des moyens adaptés et une coordination efficace entre l’État, les entreprises et les collectivités territoriales. Ce texte va plus loin que la transposition, puisqu’il élargit, dans son article 62, le champ d’application de la résilience opérationnelle numérique au secteur financier.

dans notre dispositif de protection. Cependant, il sera impératif de lui donner les moyens nécessaires à la réalisation de ses missions. Si nous pouvons nous en réjouir, nous devons cependant nous assurer que les obligations imposées par ce texte ne deviennent pas un fardeau insurmontable pour nos entreprises et nos administrations. La cybersécurité doit être perçue non pas comme une contrainte, mais comme un investissement stratégique pour garantir la pérennité de notre économie et la sécurité de nos concitoyens. Il nous faudra donc veiller à accompagner les acteurs concernés, notamment les petites et moyennes entreprises, qui sont les plus fragiles face à ce danger, dans la mise en conformité avec ces nouvelles exigences. L’État doit jouer son rôle en assurant une coordination efficace et en mettant à disposition les ressources nécessaires, mais les entreprises et les collectivités locales ont également un rôle essentiel à jouer. Ce projet de loi représente une avancée majeure, mais il ne doit être qu’une étape. C’est avec cette ambition que je vous invite, mes chers collègues, à le soutenir et à poursuivre ensemble notre engagement

marqué par la montée en puissance du numérique et de l’intelligence artificielle. Malheureusement, on constate un recours de plus en plus désinhibé de certains pays bien identifiés à des stratégies d’influence et à des actes malveillants. Dans ce contexte, la sécurité de nos infrastructures n’est plus une option elle est tout simplement vitale. Le texte est néanmoins source de préoccupation pour les plus petites entités, qui peuvent être d’une importance critique pour notre souveraineté. Je pense en particulier aux entreprises qui forment notre base industrielle et technologique de défense, aux côtés des grands groupes industriels aux côtés des grands groupes industriels dont elles sont souvent les sous traitants et les fournisseurs. Ces entreprises ne disposent pas toutes des ressources financières, humaines et organisationnelles pour satisfaire aux nouvelles normes qui vont entrer en vigueur avec cette loi. Une étude menée par la direction 300 entreprises a d’ailleurs révélé un niveau de maturité cyber très faible. Le groupe socialiste déposera plusieurs amendements afin de fixer un calendrier d’application progressif et différencié des mesures de contrôle en fonction du niveau de préparation des entités concernées,

Vous l’aurez compris, nous soutenons la mise en place de toutes les mesures qui peuvent assurer la protection de nos entreprises, mais souhaitons les accompagner au mieux pour préserver leur compétitivité. La parole

de l’intelligence artificielle et de la robotique. Madame la ministre, il est impératif de protéger les entreprises françaises des risques d’appropriation par des acteurs

introduite en commission. Le Gouvernement propose de revenir à la rédaction initiale de l’alinéa 7 de l’article 1. Notre commission a en effet adopté un amendement visant à préciser le champ des activités d’importance vitale en reprenant le texte de la directive, qui retenait des notions de santé publique et d’environnement. Pour autant, comme l’indique le Gouvernement, ce champ ne recoupe pas tout à fait celui des services essentiels de la directive REC. Aussi, je suis favorable à cet amendement.

explicitement la nécessité pour l’opérateur d’adopter des mesures efficaces qui lui permettent de résister face aux conséquences d’un incident. Il nous semble plus logique de revenir à la version initiale du texte.

souhaitons que l’autorité administrative recueille les observations d’un opérateur avant de le désigner en tant qu’opérateur d’importance vitale (OIV). L’objectif est simple : garantir que cette désignation, qui a nécessairement des conséquences importantes importantes en matière de coût et d’organisation, soit réfléchie et adaptée aux réalités de chaque acteur concerné. Cette consultation permettra de prendre en considération des facteurs essentiels, tels que la taille de l’opérateur, qui va de la TPE au grand groupe, les risques spécifiques à son secteur et sa capacité à assurer la résilience de ses infrastructures. Cette procédure figure d’ores et déjà dans le code de la défense, aux termes duquel, lorsque l’autorité administrative notifie à l’opérateur son intention de le désigner comme OIV, celui ci dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses observations. Nous proposons de consacrer ce principe dans la loi, compte tenu des implications que la désignation en tant qu’OIV entraîne. Il s’agit d’une simple mesure de bon sens que je vous invite à soutenir, mes chers

observations. Cette possibilité est déjà prévue par l’article R. 1332 3 du code de la défense. Néanmoins, la rédaction de cet amendement nous pose problème. En effet, dans l’hypothèse où l’opérateur ne produirait aucune observation,

Le sujet qui nous occupe aujourd’hui est d’importance critique pour la cybersécurité de notre nation. Cependant, il nous faut l’aborder avec un certain pragmatisme et ne pas surtransposer ; or la question de la sous traitance ne fait pas partie de la directive REC, laquelle mentionne seulement les chaînes d’approvisionnement. Il nous semble donc nécessaire de revenir au texte

par la commission spéciale me semblait pourtant renforcer le dispositif de résilience des activités d’importance vitale, la chaîne de sous traitance pouvant constituer une source de vulnérabilité à part entière. Pour autant, je suis sensible aux arguments du Gouvernement, qui considère que l’extension de l’analyse des dépendances aux sous traitants pourrait se traduire par une charge supplémentaire pour les opérateurs. Aussi, dans la

au sens de la directive REC. La rédaction actuelle de l’article 1 ne distingue pas, dans le plan particulier de résilience, ce qui relève des équipements de ce qui dépend des dispositions et des procédures mises en œuvre par l’opérateur. le plan particulier de résilience se doit de mentionner, au delà des seules procédures propres à assurer la protection et la résilience de ces points d’importance vitale,

peuvent demander l’avis de l’autorité administrative compétente, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Il convient d’assortir ce décret

et au traitement automatisé des données personnelles, ce qui soulève des questions quant à la protection de ces dernières. L’objectif de cet amendement est donc de garantir un juste équilibre entre la sécurité des infrastructures critiques

après avis de la Cnil. En effet, ces enquêtes pourront impliquer notamment la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, ainsi que le recours à des traitements automatisés de données personnelles, données de nature sensible dont le traitement doit être défini avec la plus grande vigilance pour garantir le respect des libertés individuelles. Face à cet élargissement des pouvoirs d’enquête, il nous a paru essentiel que la mise en œuvre de ces procédures soit éclairée et encadrée par l’expertise de la Cnil.

nous prévoyons un plan national permettant de structurer cet accompagnement pendant une durée de cinq ans en prévoyant divers dispositifs, notamment : l’identification précise des compétences nécessaires ; la mise en place d’un soutien technique concret pour aider les entités à évaluer leurs risques ; la définition des mécanismes d’aide financière ciblés pour les PME TPE et les collectivités territoriales ; la clarification du rôle et du financement des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique territoriaux ; et la réalisation d’un bilan de la mise en œuvre de la directive deux ans après sa promulgation, afin d’évaluer les difficultés rencontrées et d’ajuster les mesures d’accompagnement en fonction des besoins constatés sur le terrain. Un accompagnement progressif nous paraît essentiel pour garantir une mise en conformité efficace et éviter d’imposer des charges disproportionnées aux plus petites structures, tout en assurant une élévation générale du niveau de cybersécurité.

Dans le contexte de la transposition de la directive NIS 2, cette stratégie devra bien sûr revenir en détail sur l’indispensable accompagnement des PME TPE et des collectivités territoriales dans leur montée en maturité cyber. C’est la raison pour laquelle

subissent de plus en plus de cyberattaques qui emportent de nombreuses conséquences : coût des réparations, interruption des services ou de l’activité pouvant avoir des conséquences graves, vol de données. Le travail de transposition des directives européennes réalisé aujourd’hui est donc crucial pour que l’ensemble des États membres de l’Union européenne disposent d’un niveau de protection efficace et harmonisé. En France, c’est l’Anssi, en première ligne dans l’application de la directive NIS 2, qui devra relever au moins deux grands défis. Le premier défi est celui de l’appropriation par les entités concernées de leurs nouvelles obligations. L’Agence devra construire un cadre de confiance avec les entreprises et les près de 1 500 collectivités territoriales concernées ; pour ces dernières, la mise en conformité nécessitera d’importants moyens humains et financiers. Le Gouvernement donc les accompagner dans le cadre des prochaines lois de finances. Cela doit faire partie de l’effort global de défense dont M. Lecornu n’a pas manqué de parler ces derniers jours. Vous l’avez rappelé, madame la ministre, la menace

européenne compétitive, susceptible de répondre à la demande qui découlera de l’application des directives. Nos entreprises fournissent des solutions fiables et imperméables aux lois extraterritoriales. Elles doivent prioritairement bénéficier de l’effet de ruissellement suscité par la loi. Il y a là un enjeu économique d’emploi, mais aussi de souveraineté. C’est la raison pour laquelle j’ai absolument tenu à préciser que les missions de l’Anssi comprennent aussi l’accompagnement et le soutien au développement de la filière cybersécurité

Fabien Gay. Il ne peut y avoir de stratégie nationale en matière de cybersécurité sans souveraineté numérique. Au vu des bouleversements mondiaux – nul besoin d’en dire plus –, on ne peut pas se résigner ou être réduit à acheter ou louer des solutions

Quel est l’avis de la commission spéciale ? La stratégie nationale en matière de cybersécurité devra avant tout se concentrer sur les moyens de protéger nos entreprises, nos administrations et nos collectivités territoriales contre les attaques cyber qui peuvent paralyser leurs services et lourdement les pénaliser, tout comme leurs utilisateurs. Il faut bien sûr encourager parallèlement le développement en France de l’écosystème des entreprises spécialisées en matière de cybersécurité, mais il ne paraît en pratique pas possible de prétendre avoir recours uniquement à des technologies françaises ou européennes. Pour ce qui relève de la souveraineté numérique,

Quel est l’avis du Gouvernement ? Monsieur le sénateur, vous mentionnez l’importance de la stratégie cyber. Je vous rejoins sur ce point. Elle a été présentée pour la première fois en 2015, réactualisée en 2018 et en 2021 ; le Président de la République a annoncé à la fin de l’année dernière

en faveur de la souveraineté numérique. Aujourd’hui, on pleure parce qu’on se rend compte, dans le nouveau contexte international, que nos dépendances technologiques sont très dangereuses.

l’amendement n° 65. Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à minuit et demi.

Leur importance est consacrée par l’article 24 du projet de loi, qui prévoit leur agrément afin de leur donner plus de poids et d’importance dans la politique de cybersécurité du pays. Il est dès lors très opportun que la stratégie nationale en matière de cybersécurité précise leur cadre d’intervention et leur déploiement dans tous les territoires, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Pour autant, l’ajout de cet alinéa ne me paraît pas indispensable. Cet

cloud localisés en Europe, financés par des capitaux européens et nationaux. Notre collègue Catherine Morin Desailly a parfaitement nos faiblesses et nos lenteurs en la matière. L’enjeu est donc bien de soutenir les acteurs européens et de défendre nos intérêts numériques et géostratégiques. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

Je vous remercie

spéciale ? Le renforcement des compétences et des formations nécessaires en matière de cybersécurité sur l’ensemble des territoires est bien sûr une priorité et devra être traité comme tel par la stratégie nationale

aurons plusieurs débats sur le contexte géopolitique international : la cybersécurité sera abordée dans ce cadre. Je n’ai pas de réponse plus précise à vous apporter sur ce dispositif particulier, mais sachez que nous avons bien en tête la nécessité de continuer à renforcer la cybersécurité.